Mes chers collègues, il va être procédé dans les conditions prévues par l'article 86 du règlement au scrutin secret pour l'élection de six juges titulaires et de six juges suppléants à la Cour de justice de la République. Ce scrutin se déroulera dans la salle des conférences et la séance ne sera pas suspendue durant les opérations de vote. Je rappelle que la majorité absolue des suffrages exprimés est requise pour être élu. Pour être valables, les bulletins ne peuvent comporter plus de six noms pour les juges titulaires et plus de six noms pour les suppléants. Le nom de chaque titulaire doit être obligatoirement assorti du nom de son suppléant. En conséquence, la radiation de l'un des deux noms, soit celui du titulaire, soit celui du suppléant, entraîne la nullité du vote pour l'autre. Une seule délégation de vote est admise par sénateur. Je remercie nos collègues Éric Bocquet et Dominique de Legge, secrétaires du Sénat, qui vont superviser ce scrutin. Les juges titulaires et les juges suppléants à la Cour de justice de la République nouvellement élus seront immédiatement appelés à prêter serment devant le Sénat. Je déclare ouvert le scrutin pour l'élection de six juges titulaires et de six juges suppléants à la Cour de justice de la République. Il sera clos dans une demi-heure. L'ordre du jour appelle la désignation des dix-huit sénateurs membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques membres de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes ; des trente-six membres de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation

En application des articles 110 et 8 du règlement du Sénat et du chapitre IV de l'instruction générale du Bureau, les listes des candidats présentés par les groupes ont été publiées. Ces candidatures seront ratifiées si la présidence ne reçoit pas d'opposition dans le délai d'une heure. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme

madame la ministre auprès du ministre de l'intérieur, mes chers collègues, nous arrivons au terme de l'élaboration d'un texte qui n'est pas sans poser un grand nombre de difficultés. nous l'avons déjà débattu et voté au mois de juillet dernier, avant qu'il ne soit modifié par l'Assemblée nationale. Il nous revient après un accord trouvé en commission mixte paritaire.

Si l'état d'urgence permet à l'État d'utiliser des dispositifs conférant une efficacité maximale à la lutte contre le terrorisme, c'est parce que ces mesures sont temporaires, temporaires, qu'elles donnent lieu à un contrôle parlementaire- elles ne peuvent être prorogées au-delà de quelques mois sans un nouveau vote du Parlement -et qu'elles sont soumises à un contrôle de proportionnalité du juge administratif. Dans le respect de ces conditions, les mesures de l'état d'urgence sont acceptables, malgré les restrictions qu'elles apportent aux libertés publiques, dont le Sénat est historiquement un défenseur, tout en ayant à coeur de donner à l'État les moyens de la lutte contre l'insécurité. À l'aune des libertés fondamentales, la loi permanente ne peut donner à l'État les mêmes pouvoirs que la loi d'exception. La loi d'exception peut déroger au droit commun ; le droit commun ne peut déroger à l'État de droit.

au point que l'État pourrait substituer à l'état d'urgence sa réplique, dans une version atténuée, pour ne pas dire dégradée Cette version, qui figure dans le texte que nous avons à approuver, présente deux caractéristiques : elle donne moins d'armes à l'État que l'état d'urgence pour lutter contre le terrorisme, mais elle est plus contestable du point de vue des libertés, à partir du moment où il s'agit de modifier le droit permanent et non de mettre en oeuvre des mesures d'exception. Madame la ministre, vous le savez mieux que quiconque, le Sénat a su prendre à plusieurs reprises l'initiative de renforcer la loi permanente pour améliorer nos moyens d'action. C'est dire que nous ne sommes nullement hostiles, par principe, à un certain durcissement de la loi répressive et à un certain renforcement des pouvoirs de l'autorité administrative. Nous l'avons fait lors de l'examen de la loi sur le renseignement. Nous l'avons fait dès le mois de février 2015, après les terribles attentats de janvier, lorsque j'ai proposé au nom de la majorité sénatoriale, au Premier ministre de l'époque, des mesures ayant une portée législative. Ces propositions sont malheureusement restées sans réponse. Nous nous sommes donc mis au travail, afin d'élaborer une proposition de loi pour renforcer la lutte contre le terrorisme, le terrorisme, déposée en décembre 2015. Après les attentats du mois de novembre 2015, le Gouvernement a annoncé un certain nombre de décisions, notamment qu'il mettait enfin en chantier une loi pour renforcer la lutte

pour que ces dispositions deviennent la loi du 3 juin 2016, suivie après l'attentat de Nice d'une nouvelle loi qui, d'un côté prorogeait l'état d'urgence, et, de l'autre, de l'autre, prévoyait l'entrée en vigueur de celles des mesures que nous avions prévues et qui n'avaient pas été adoptées dans la loi du 3 juin. Ainsi, l'ensemble de l'arsenal renforçant la lutte contre le terrorisme au cours des dernières années résulte en réalité de propositions du Sénat de la République. C'est dire que, sur le chapitre de la lutte contre le terrorisme, nous pouvons témoigner, face à l'opinion publique, que le Sénat a à coeur de renforcer les moyens de la sécurité. Nous ne pouvons donc par principe récuser aujourd'hui l'idée d'un nouveau renforcement des moyens de l'État proposé dans ce texte, bien au contraire. Ce que nous récusons, c'est seulement l'idée que celui-ci pourrait se substituer à l'état d'urgence

Rapporteur du projet de loi en première lecture, notre éminent collègue Michel Mercier, avec sa longue expérience de ces questions et son discernement de grand juriste et d'ancien garde des sceaux, s'était évertué avec efficacité à sauver ce texte sécuritaire en cantonnant les restrictions qu'il implique pour les libertés individuelles et les libertés publiques au strict nécessaire, afin d'éviter le risque d'une censure constitutionnelle. Tel est bien l'exercice auquel nous devons nous soumettre : aller le plus loin possible dans le renforcement de notre arsenal sécuritaire de droit commun, sans franchir la ligne rouge à partir de laquelle nos libertés seraient durablement atteintes. Il s'agit de donner sa pleine efficacité à la lutte contre le terrorisme, dans le respect de notre État de droit et de nos traditions républicaines. C'est une gageure Le rapporteur que je suis, au pied levé, n'est pas en mesure d'apporter la garantie que toutes les dispositions du texte du Gouvernement, même amendé par le Sénat et rediscuté en commission mixte paritaire, pourront franchir le cap d'un examen éventuel par le Conseil constitutionnel. Pourtant, nous nous sommes donné du mal ! Nous avons inventé au mois de juillet dernier une « clause d'autodestruction

tomberont d'elles-mêmes au bout d'un certain délai. Si le Gouvernement estime à ce moment-là qu'il est nécessaire de les reconduire, il devra revenir devant nous. C'est ainsi que nous donnons un caractère temporaire à la loi permanente, même si cette temporalité est plus longue que celle que nous avons l'habitude d'accepter quand il s'agit de l'état d'urgence. La temporalité est plus longue, mais les mesures sont moins restrictives pour les libertés. Sans doute le Conseil constitutionnel pourrait-il accepter un tel équilibre. Toutefois,

de sécurité à l'intérieur desquels on n'entre pas sans montrer patte blanche, sans être invité à subir des fouilles et à prouver son identité, toutes ces mesures

-de la transmission au Parlement de tous les éléments factuels d'information sur la mise en oeuvre de ces mesures, sur la manière dont le juge les aura appréciées et sur leur utilité pour la lutte contre le terrorisme. Le Sénat a par ailleurs encadré la mise en oeuvre de chacune des principales mesures prévues par le projet de loi. Il a renforcé le pouvoir du juge

Je puis néanmoins assurer que, si le Gouvernement persiste dans son intention de ne pas nous demander la prorogation de l'état d'urgence, le dispositif que nous aurons adopté aujourd'hui nous permettra à la fois de renforcer nos armes dans la lutte contre le terrorisme, sans pour autant mettre en péril nos libertés.

Madame la présidente, monsieur le rapporteur et président de la commission des lois, mesdames, messieurs les sénateurs, la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme est parvenue à un accord, et le Gouvernement s'en réjouit. En effet, je me félicite que les représentants des deux assemblées soient parvenus à un texte commun sur un sujet aussi important. Sur ces questions essentielles que constituent la lutte contre le terrorisme et les moyens que nous mettons en oeuvre pour assurer notre sécurité, nos concitoyens ne comprendraient pas que nous ne sachions pas nous rassembler et faire preuve d'unité nationale.

Avec cet accord en commission mixte paritaire, qui fait suite à l'approbation à de larges majorités du texte dans les deux assemblées parlementaires- 229 voix pour au Sénat, 415 voix pour à l'Assemblée nationale -, nous avons, je crois, été collectivement à la hauteur de cet enjeu majeur. Bien entendu, je tiens à remercier l'ensemble des sénateurs qui ont participé de manière active aux travaux sur ce texte et ont contribué à son enrichissement et à son amélioration. Je pense tout d'abord à M. Philippe Bas, président de votre commission des lois, qui a repris, après le renouvellement sénatorial du mois dernier,

de la commission, le travail effectué par Michel Mercier en première lecture sur ce projet de loi et, de manière plus générale, saluer son investissement et sa contribution déterminante, au cours des trois dernières années,

Qu'il me soit enfin permis de saluer l'ouverture d'esprit et le sens du compromis dont ont su faire preuve tous les membres de la commission mixte paritaire pour parvenir à cet accord. À force de discussions, de pédagogie au fil des débats devant les deux assemblées parlementaires, au cours desquels nous avons étudié des centaines d'amendements, nous avons fait en sorte de converger. Oui, c'est vrai, ce texte a été fortement discuté et débattu. Son adoption n'allait pas de soi, tant il pouvait paraître inapproprié, pour ne pas dire inenvisageable, de sortir de l'état d'urgence compte tenu du maintien, sur notre territoire, d'une menace terroriste à un niveau extrêmement élevé. Nous y avons été à nouveau collectivement confrontés, malheureusement, le 1 octobre dernier, avec cet acte lâche et barbare qui a enlevé la vie à deux jeunes filles, Laura et Maurane, âgées qui se trouvaient au mauvais endroit au mauvais moment. Nous l'avons également vu avec les bonbonnes de gaz découvertes dans le hall d'un immeuble du XVI arrondissement de Paris, ou encore avec le projet d'attentat qui se fomentait dans un établissement pénitentiaire de la région parisienne. Dans un tel contexte, le Gouvernement, nos forces de sécurité intérieure nos services de renseignement, dont je veux saluer le dévouement, le professionnalisme et l'efficacité, ont une obligation et une seule : tout faire pour entraver, dans le respect de l'État de droit, les individus qui présentent une menace pour notre sécurité tout faire pour garantir la sécurité de nos concitoyens. Je veux ainsi rappeler que, depuis le début de l'année 2017, ce sont cinq attaques terroristes qui ont été entreprises, ayant coûté la vie à trois personnes, qui ont échoué et treize qui ont été déjouées par l'action de nos services. Je veux à cet égard préciser que les mesures de police administrative prises par les autorités administratives ont joué, pour nombre de ces attentats entravés, un rôle absolument déterminant. Comme cela a été souligné à de nombreuses reprises lors des débats parlementaires, la menace terroriste évolue, change de nature hier orchestrée depuis les terres contrôlées par Daesh, elle est aujourd'hui endogène, oeuvre d'individus qui, radicalisés, utilisent tous les moyens pour agir. Surtout, et ce constat n'est pas récent, elle est devenue durable, malgré les importants revers militaires que subit sur le terrain le prétendu État islamique. Qu'était-il possible de faire dans un tel contexte ?

Cette option a été vigoureusement défendue par le groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, lequel a accusé le Gouvernement, tout au long des débats, de désarmer notre pays face à la menace terroriste.

peut-on raisonnablement demeurer encore dans l'état d'urgence, alors que nous y vivons désormais depuis plus de deux ans ? Le Gouvernement ne le pense pas et fait sienne la formule du Conseil d'État, monsieur le président selon laquelle « l'état d'urgence est un régime de pouvoirs exceptionnels ayant des effets qui, dans un État de droit, sont par nature limités dans le temps et dans l'espace Face à une menace devenue durable, il nous faut avoir recours à des instruments ayant vocation à y répondre de façon permanente. C'est cette voie que le Gouvernement a entendu privilégier en partant du constat qu'il convenait, après deux années d'application de ce régime juridique exceptionnel, de sortir de l'état d'urgence tout en réfléchissant aux outils pouvant alors faire défaut à nos services pour lutter contre la menace terroriste. Ce texte, mesdames, messieurs les sénateurs, est exclusivement destiné à lutter contre le terrorisme pour ce qui concerne ses quatre premiers articles, qui ont été les plus débattus. Contrairement aux mesures de police administrative de l'état d'urgence, ces nouveaux outils ne permettent pas de lutter contre des menaces à la sécurité et à l'ordre publics, mais sont prévus « aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme Certes, nous n'avons pas la prétention d'affirmer que ce texte nous permettra d'éradiquer le péril terroriste et d'éviter les attentats. Qui pourrait le prétendre ? Au demeurant, les attentats commis, échoués ou entravés en 2017 démontrent à eux seuls que l'état d'urgence ne constitue pas non plus un bouclier contre le terrorisme. Toutefois, le Gouvernement a une certitude. Au travers de ce texte que vous vous apprêtez à adopter, nous mettons de notre côté toutes les chances de prévenir en amont la commission d'actes de terrorisme, en permettant de prévenir le processus de radicalisation avec la fermeture des lieux de culte où seraient diffusées des idées de haine, de violence, incitant à la commission d'actes terroristes, mais aussi en donnant à nos forces de sécurité la possibilité de prévenir des attentats imminents, par la surveillance d'individus, voire par des visites à leur domicile, quand tout laisse à penser qu'ils sont sur le point de passer à l'acte. Mesdames, messieurs les sénateurs, je ne vais pas rappeler ici l'ensemble des articles que contient le projet de loi et je ne présenterai pas plus de manière exhaustive les termes de l'accord conclu en commission mixte paritaire, puisque le président Philippe Bas vient d'en rappeler l'essentiel. Je souhaiterais simplement dire un mot des principales dispositions renforçant les outils de lutte contre le terrorisme qui seront demain à la disposition de nos forces de sécurité. Je me réjouis tout d'abord de la rédaction consensuelle qui a été retenue pour l'article 1 relatif aux périmètres de protection, qui sera de nature à permettre aux Français d'assister à de grands événements culturels, récréatifs ou sportifs, tout en donnant aux autorités de police la possibilité d'en assurer la sécurité. Les terroristes ne nous feront pas renoncer à notre mode de vie. Nous ne leur céderons rien sur ce plan. Concernant l'article 2 relatif à la fermeture des lieux de culte, la formulation retenue par la commission mixte paritaire est particulièrement satisfaisante. Il était pour le Gouvernement essentiel, pour garantir l'efficacité de notre action, de conserver les notions les notions de diffusion d'« idées » et de « théories », ainsi que les mentions d'incitation à la « haine » et à la « discrimination », pour motiver la fermeture d'un lieu de culte. Vous savez du reste que le Gouvernement a agi avec discernement en la matière pendant l'état d'urgence, puisque ce sont dix-huit lieux de culte qui ont été fermés depuis le 14 novembre 2015, seuls dix d'entre eux le demeurant à l'heure actuelle. Demain, avec la nouvelle loi, nous entendons continuer à agir dans le même état d'esprit. Sur l'article 3, qui comprend les mesures de surveillance individuelle, la commission mixte paritaire est parvenue à l'établissement d'un texte équilibré. Le Gouvernement était attaché à la possibilité d'imposer un pointage quotidien auprès des services de police ou de gendarmerie, et je veux remercier le Sénat de s'être rallié à notre opinion sur ce point. D'une manière générale, la navette parlementaire a permis de renforcer les garanties qui s'attachent à ce dispositif, dont l'application ne pourra excéder une année et dont chaque renouvellement, tous les trois ou six mois selon les obligations, sera assorti d'une procédure permettant aux personnes concernées de saisir le juge. Sur l'article 4, relatif aux visites et saisies, le Gouvernement relève également le caractère équilibré de la rédaction approuvée.

Nous aurons donc l'occasion d'évaluer, avant le 31 décembre 2020, l'ensemble des quatre premiers articles du présent texte. Enfin, j'évoquerai l'article 10, qui porte sur les contrôles d'identité aux abords des points de passage aux frontières

Cette modification renforce le caractère proportionné des mesures prévues, tout en permettant des contrôles aux alentours des points de passage aux frontières les plus sensibles.

nous sortons de l'état d'urgence, nous maintiendrons, grâce à ce texte de loi, un haut niveau de protection contre le terrorisme. Il n'est pas question de nous désarmer face à un ennemi qui continuera à tenter de porter des coups à tous nos pays durant une longue période.

afin de garantir à nos concitoyens le niveau le plus élevé possible de sécurité. Mes chers heures et deux minutes. Je déclare clos le scrutin pour l'élection de six juges titulaires et de six juges suppléants à la Cour de justice de la République.

madame la ministre auprès du ministre de l'intérieur, mes chers collègues,

la nécessaire sortie de l'état d'urgence et la pertinence d'inscrire les mesures utiles de l'état d'urgence dans le droit commun. Premièrement, j'insisterai sur la nécessaire sortie de l'état d'urgence.

nous le savons tous. Il nous restait à sortir de l'état d'urgence sans désarmer l'État de droit. La commande passée par le Président de la République et par le Gouvernement devait aboutir à l'assimilation politique et juridique des dispositions pertinentes issues de l'état d'urgence dans notre droit commun de la lutte antiterroriste. Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui atteint cet objectif. Nous revenons à une situation classique, hiérarchisée, avec un droit commun, la possibilité pour le Gouvernement de recourir à l'état d'urgence en lien avec le Parlement, enfin, au-dessus, l'état de siège. Deuxièmement, j'évoquerai la pertinence de conserver les mesures utiles de l'état d'urgence dans le droit commun. La commission mixte paritaire a validé sur plusieurs points

puisque cette clause ouvre la possibilité au législateur de revenir sur le sujet, de proroger, de pérenniser et de réécrire les dispositions en vigueur en fonction de l'évolution des menaces dans le temps. Nous estimons être parvenus au terme du processus législatif de lutte contre le terrorisme avec un véritable arsenal juridique, puisque, au cours des quatre dernières années, huit lois ont été adoptées. Nous sommes aussi arrivés aux limites de la créativité juridique acceptable, aux limites de l'équilibre entre sécurité publique et libertés publiques, avec un droit administratif qui a évolué vers la sanction et un droit pénal qui intervient très en amont du passage à l'acte et frise ainsi la notion de prévention.

Deuxièmement, comment traiter les djihadistes déjà condamnés, incarcérés, mais qui finiront par être libérés ? Autrement dit, que faire de personnes déjà radicalisées, qui le seront probablement d'autant plus à leur sortie de prison, et qui pourraient avoir pour seul désir de se transformer en bombes humaines

il faut sans doute pouvoir affirmer : « Oui, je quitte l'état d'urgence, mais je mets l'état d'urgence dans le droit commun. » Ainsi, on aboutit à ce texte de loi, qui doit permettre de sortir de l'état d'urgence tout en y restant un peu. Voilà comment les faits se sont enchaînés.

nous dit-on, cesseront automatiquement le 31 décembre 2020- c'est le sens de l'article 4 A -, à cette nuance près

mi-administrative, mi-judiciaire. Le juge des libertés du tribunal de grande instance de Paris doit l'autoriser, mais c'est l'administration qui la met en oeuvre. Par

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur et président de la commission des lois, mes chers collègues, je tiens tout d'abord, du haut de cette tribune, à partager avec vous une pensée pour les victimes du terrorisme et pour leurs proches, mais aussi à rendre un hommage appuyé aux services de police, de gendarmerie, de renseignement et de défense, qui concourent jour et nuit à notre sécurité en prenant de grands risques. J'ai pu apprécier le sérieux, l'application et l'abnégation de tous ces personnels lorsque j'étais rapporteur du budget des sécurités. L'état d'urgence est par nature limité dans l'espace et dans le temps. Il doit rester temporaire et exceptionnel. Parce que voici vingt-trois mois que l'état d'urgence est entré en vigueur, la question de son maintien se pose actuellement de façon accrue. En l'espace de deux ans, de nombreuses mesures ont été prises. Ainsi, nous sommes mieux préparés à faire face au risque terroriste qu'à l'époque du Bataclan. Notre connaissance de la menace et nos capacités d'enquête se sont améliorées. Les effectifs de nos services de sécurité ont été renforcés. de proroger l'état d'urgence indéfiniment, il ne faut pas non plus revenir à la situation antérieure à l'état d'urgence. Il convient donc de prendre des dispositions qui visent à protéger les citoyens tout en garantissant leurs libertés des dispositions qui apportent une réponse durable à une menace devenue durable en adaptant notre droit commun. Et c'est une constante du Sénat, loin des pulsions médiatiques et de l'actualité brûlante, que de garantir ces libertés. Les mesures de ce projet de loi ne visent que le seul terrorisme et ne sont pas prises pour des motifs ayant trait à l'ordre public, comme dans le cadre de l'état d'urgence. Les principales d'entre elles sont au nombre de quatre. Inspirées de l'état d'urgence, elles sont mises, dorénavant, à la disposition de nos services de sécurité. Ces quatre outils sont les périmètres de protection ; la fermeture administrative des lieux de culte ; les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance ; enfin, les visites domiciliaires et saisies. L'article 1 vise ainsi à permettre l'institution de périmètres de protection, sans lesquels il serait désormais impossible d'organiser de grands rassemblements. Il est particulièrement important de toujours disposer des instruments permettant d'organiser des manifestations de cette ampleur tout en garantissant la sécurité de tous ceux qui y assistent. L'article 2 prévoit la possibilité pour le représentant de l'État de prononcer la fermeture des lieux de culte. Par cette disposition, les préfets ou le préfet de police doivent pouvoir prévenir la menace en fermant les lieux où la radicalisation serait prônée et où serait pratiquée l'incitation au passage à l'acte terroriste. L'article 3, quant à lui, concerne la création, sur décision du ministre de l'intérieur, d'un régime de surveillance individuelle. Enfin, le quatrième point emblématique est le régime des visites et saisies à domicile. La commission mixte paritaire a élargi la clause d'autodestruction introduite par le Sénat en première lecture à l'ensemble des nouveaux outils mis à disposition des autorités administratives pour prévenir la commission des actes de terrorisme. Ces quatre mesures revêtiront donc un caractère expérimental. Elles prendront fin au 31 décembre 2020 et seront soumises à un contrôle renforcé du Parlement. la commission mixte paritaire a supprimé l'obligation, pour une personne soumise à une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, de déclarer les numéros d'abonnement et les identifiants techniques de l'ensemble de ses moyens de communication électronique. Cette mesure paraissait manifestement contraire aux droits fondamentaux, dont le respect est garanti par le Conseil constitutionnel. Indéniablement, l'ensemble de ces outils présente une utilité opérationnelle, indispensable pour lutter efficacement contre le terrorisme. Ce projet de loi constitue un juste équilibre entre l'impératif de protection de l'ordre public et la préservation des libertés individuelles. Nous savons que le gouvernement est animé, comme nous tous d'ailleurs dans cet hémicycle, par un esprit de responsabilité qui conduit à mieux protéger nos concitoyens. En effet, la France est la cible privilégiée de ces barbares, parce qu'elle est tout ce qu'ils veulent détruire : le pays des libertés, le pays des Lumières. Madame la ministre, mes chers collègues, ce texte est équilibré et responsable. Il répond à l'inquiétude légitime de nos concitoyens, et c'est bien de cet équilibre que la France a besoin pour répondre à ceux qui menacent notre modèle démocratique et nos valeurs républicaines

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur et président de la commission des lois, mes chers collègues, à ce stade des discussions, après l'obtention de l'accord en commission mixte paritaire, le vote d'aujourd'hui nous met est-il préférable d'inscrire les dispositions de la loi du 3 avril 1955 dans le droit commun ou de laisser vivre le régime de l'état d'urgence au gré de reconductions illimitées ? Il est à présent certain que le Gouvernement ne prendra pas la responsabilité de lever l'état d'urgence sans avoir obtenu la faculté permanente, pour l'autorité administrative, d'ordonner des perquisitions, des assignations à résidence ou des fermetures de lieux de culte à des fins de lutte contre le terrorisme. Il est également certain que le Parlement ne prendra pas la responsabilité de voter contre un projet de loi de prorogation sans que lui soient apportés les signes d'un affaiblissement durable de la menace terroriste. Il est enfin certain que seul le Gouvernement est en mesure d'évaluer l'ampleur réelle de la menace et la faculté relative pour nos services de sécurité d'y faire face, pour des raisons évidentes de confidentialité.

abrogation improbable », est de donner au Gouvernement la capacité d'agir selon sa volonté. Toutefois, cette capacité va de pair avec la responsabilité de la mise en oeuvre de mesures qu'il devra assumer pleinement. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, notre soutien n'est pas exempt de réserves. Vous connaissez l'attachement des membres du RDSE à la protection des libertés et à son corollaire, la garantie offerte par le contrôle de l'autorité judiciaire sur les actes de l'administration. L'une et l'autre sont mises à mal par la version de compromis proposée par la commission mixte paritaire, malgré les efforts de notre rapporteur pour défendre les garde-fous introduits par le Sénat.

la liberté de mener une vie familiale sereine. Ces mesures devront donc rester exceptionnelles et strictement proportionnées aux besoins de la lutte contre le terrorisme. Nous veillerons à ce qu'elles ne soient pas détournées à des fins plus larges de protection de l'ordre public. La systématisation du recours à des mesures administratives pour lutter contre le terrorisme place le juge judiciaire en retrait : au titre de dispositions attentatoires aux libertés, le contrôle exercé par le juge administratif est moins satisfaisant pour les administrés : ces derniers ne peuvent recourir à lui qu'. Cette évolution risque également de placer le juge administratif en difficulté, tant la matière terroriste lui est peu familière, tant ses moyens d'instruction sont réduits. dans la pratique, son contrôle se borne à constater l'existence d'une note blanche dont les éléments justifient la décision prise.

Nous savons que leurs exigences déontologiques seront à la hauteur du défi. En outre, ces dispositions s'ajouteront aux nombreuses mesures que le Parlement a adoptées depuis 2015 et qui ont permis d'étendre considérablement les moyens légaux de renseignement et de protection. Il me semble que nous sommes allés au bout de ce qu'autorisent notre droit constitutionnel et nos engagements internationaux pour permettre à nos forces de l'ordre d'agir. Aller plus loin, en donnant le droit à toutes les institutions qui le réclament de constituer leurs propres services de sécurité ou d'incarcérer préventivement l'ensemble des individus fichés S, serait mettre le doigt dans un engrenage qui nous éloignerait progressivement de notre identité constitutionnelle.

notre désir farouche de neutraliser les dessins funestes du terrorisme doit être traité indépendamment de tous les autres sujets, afin de gagner en efficacité et d'éviter de déclencher des débats douloureux sur l'existence d'amalgames. C'est pourquoi nous regrettons le maintien de l'article 10, qui aurait davantage sa place dans une loi consacrée à la lutte contre l'immigration irrégulière. Malgré toutes ces réserves, la suppression de la possibilité de collecter les identifiants et les mots de passe de personnes suspectées d'être en lien avec des organisations terroristes et plus encore l'instauration d'une clause d'autodestruction en 2020 nous apparaissent comme des garanties bienvenues. Nous voterons donc en majorité en faveur de l'adoption, conformément à notre position en première lecture et afin de donner à ce nouveau gouvernement la possibilité d'assumer sa politique. Néanmoins, ce choix ne nous empêchera pas de réfléchir, à l'avenir, à l'effet cliquet des lois temporaires.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, notre assemblée se trouve devant une interrogation politique douloureuse, comme nous en rencontrons parfois. Face à un péril resté intense et que nous sommes obligés de juger durable, comment pouvons-nous adapter notre législation aux enjeux de sécurité qui persistent ? Le Président de la République a annoncé le choix de mettre fin à l'état d'urgence. C'est un choix que beaucoup peuvent partager, puisque l'état d'urgence est caractérisé par son caractère exceptionnel et temporaire.

par l'état d'urgence et d'en tirer les leçons, de manière à faire face à ce péril que nous savons durable. Dans le projet de loi que nous examinons, deux mesures sont en réalité des mesures de police administrative établies, mais clarifiées par la loi : la fermeture de lieux de culte et le périmètre de protection. Ces mesures-là ne sont pas spécifiquement

pour faire obstacle aux préparatifs d'actions terroristes : la limitation des mouvements de personnes sous le contrôle du juge administratif et la visite et saisie domiciliaire avec l'accord du juge des libertés et de la détention. Ces dispositions sont en effet plus intrusives.

critiquant et mettant fin à des actes de police administrative pendant l'état d'urgence. J'ajoute, pour répondre à la collègue qui m'a précédé, qu'en complétant son information elle pourrait être assurée de la capacité technique du juge administratif à faire face à ces questions, notamment depuis qu'a été créée une formation spécifique au sein du Conseil d'État.

Voilà qui nous conduit à considérer que l'équilibre et la pertinence de ces mesures nouvelles sont satisfaisants et que nous devons les soutenir. L'enjeu, en effet, c'est l'efficacité de la prévention, laquelle va rester indispensable. Le risque d'attentat, les tentatives, les préparatifs, les mouvements transfrontaliers avec les retours de la zone de combat continueront à faire apparaître des risques imminents face auxquels il faut des mesures adaptées.

La limitation des mouvements de l'intéressé, évidemment sous le contrôle du juge et pour une durée limitée, est un moyen de soulager la pression sur les services actifs de renseignement et, par conséquent, de leur permettre de mieux cibler leurs actions. Les capacités sont donc mieux utilisées et nous adaptons les outils de la police administrative à une menace qui est maintenant mieux connue. Chaque groupe, chaque sénateur, est placé face à ses responsabilités dans ce choix. avons le devoir impérieux de montrer notre détermination à lutter contre un péril qui menace la République et ses citoyens au quotidien et d'exprimer notre vigilance dans la protection des libertés individuelles. À l'issue de cette appréciation, notre groupe approuve le projet de loi, comme, je crois, une large majorité d'entre nous.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, il y a tout juste trois mois, j'intervenais ici même pour présenter une motion du groupe communiste républicain et citoyen tendant à opposer la question préalable afin que soit rejeté l'ensemble de ce projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. donc pas surpris qu'aujourd'hui notre position sur le texte issu de la commission mixte paritaire soit sensiblement la même.

lequel estime que le projet de loi final est équilibré entre mesures de sécurité et maintien des valeurs de liberté. Madame la ministre, le le Gouvernement a été hermétique aux voix extérieures des associations de protection des libertés publiques et autres syndicats vertement opposés à l'état d'urgence, mais aussi aussi du Défenseur des droits, Jacques Toubon, ou encore des experts de l'ONU. Il a été également hermétique aux voix des parlementaires opposés depuis bientôt deux ans à ce déferlement de mesures administratives toujours plus sécuritaires. Plus encore, il n'a pris en compte les maigres améliorations proposées par la commission des lois du Sénat qu'en dernier recours. L'obligation pour une personne soumise à une mesure individuelle de surveillance de déclarer les numéros d'abonnement et les identifiants techniques de ses moyens de communication électronique, que d'ailleurs la mesure la plus inconstitutionnelle du texte. En revanche, la demande des sénateurs, qui souhaitaient que le juge des libertés et de la détention donne son accord pour la retenue sur place des personnes dont le domicile est perquisitionné, a été rejetée. Finalement,

Cette question mérite pourtant mieux que cela, au lendemain d'un renouvellement présidentiel et législatif. En juillet, nous demandions l'organisation en urgence d'un débat public sur les politiques à mener pour lutter contre le terrorisme. Quand allons-nous enfin comprendre que le terrorisme appelle la prévention, bien davantage que la répression ? Qu'en est-il dans le texte qui nous est soumis ? Un seul mode opératoire est à l'oeuvre : toujours plus de répression, pas une ligne sur la prévention. Je vous le dis solennellement, madame la ministre : le terrorisme n'est pas de ces menaces que le droit peut définitivement éradiquer. Elle a raison. il échappe aux règles de l'État de droit. C'est pourquoi celui-ci n'aurait pas dû faiblir et devrait se donner les moyens de l'éradiquer autrement, en allant aux sources de sa formation, aux racines du mal. Les propositions faites à l'Assemblée nationale pour lutter contre le financement du terrorisme n'ont pas été retenues par le Gouvernement, nous le déplorons amèrement. Je le dis pour la énième fois le terrorisme se nourrit de la guerre du pétrole et du trafic d'armes. Il faut enfin dénoncer le rôle trouble des puissances régionales comme la Turquie, l'Arabie Saoudite et le Qatar, mais aussi le rôle scandaleux de certaines entreprises françaises, telles que le cimentier Lafarge. Nous le disons depuis le Congrès de Versailles du 16 novembre 2015, il faut rapidement repenser les choses et cesser d'agir en ordre dispersé. Une large coalition internationale sous mandat de l'ONU doit être mise en place, avec, au-delà du combat contre Daech, l'ambition de reconstruire les régions concernées, d'établir une paix durable et ainsi de permettre le retour de milliers de réfugiés. Sans cette perspective, pas d'issue au terrorisme. Sur le plan national, enfin, il faut refonder le vivre ensemble. D'un côté, l'accent doit être mis sur les politiques publiques de la culture et de l'éducation, le tissu associatif doit être renforcé,

contre toute forme de radicalisation en récupérant les renseignements à la source. En ce sens- vous le savez, monsieur Grosdidier -, nous sommes à l'initiative d'une proposition de loi visant à rétablir, voire à réhabiliter, la police de proximité, que nous soumettrons à l'examen de notre assemblée avant la fin de l'année. Mes chers collègues, l'heure est grave. À l'issue de cette séance, des modifications législatives d'ampleur seront définitivement adoptées. Des mesures d'exception, telles que la possibilité pour l'autorité administrative de décider de l'instauration d'un périmètre de sécurité, de la fermeture de lieux de culte, de perquisitions administratives et d'assignations à résidence, seront gravées dans notre droit commun. En votant une énième fois contre ces dispositions, contre cette dernière mouture du projet de loi, nous refusons de choisir, en toute responsabilité, de répondre à la terreur par la peur et à la menace sur nos libertés par moins de liberté. Nous resterons extrêmement vigilants quant aux applications, que nous savons déjà néfastes, de ces mesures.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il y a tout juste trois mois, jour pour jour, nous évoquions ici la pilule empoisonnée du terrorisme.

à la voiture bélier contre les militaires de l'opération Sentinelle à Levallois-Perret, le 9 août, de l'attaque au couteau dans une station de métro à Paris, le 15 septembre, et de l'attentat de la gare Saint-Charles à Marseille, le 1 octobre. Dans le même temps, ainsi que nous l'avons appris très récemment, plusieurs attentats ont été déjoués grâce aux missions ciblées et continues de nos forces de renseignement, que je tiens, en votre nom, à saluer tout particulièrement. Bien Bien sûr, l'état d'urgence a vocation à rester exceptionnel et temporaire, car il est justifié par la persistance d'un péril imminent au caractère diffus et violent. Le Gouvernement, madame la ministre, ne semble pas considérer que les conditions sont aujourd'hui réunies pour proroger de nouveau l'état d'urgence décrété au lendemain de l'attentat du Bataclan.

sont propres : le droit commun ne peut pas déroger, par définition, au principe auquel nous sommes attachés, celui de la liberté individuelle et des libertés publiques. Il faut donc que ce droit commun, aussi exceptionnel soit-il, soit cadré

Notre groupe a d'ailleurs eu une grande part dans ces évolutions, notamment à l'occasion du vote de la loi du 3 juin 2016, laquelle reprenait, pour l'essentiel, la proposition de loi que M. Philippe Bas avait déposée dès le mois de février de la même année. Nous tenions effectivement à apporter des outils juridiques et techniques permettant de répondre au manque manifeste de moyens et de procédures qui avait été constaté après les attentats de 2015.

le délit d'entrave au blocage des sites incitant à la commission d'actes terroristes et le délit de consultation habituelle de tels sites. Nous avons assuré l'exécution plus rigoureuse des peines en allongeant la période de sûreté de vingt-deux Nous avons amélioré la détection et la prise en charge de la radicalisation en imposant le suivi socio-judiciaire. Nous avons renforcé l'efficacité des investigations judiciaires en adaptant les techniques d'enquête existantes. Nous avons augmenté les pouvoirs de police administrative et du parquet en élargissant les possibilités de perquisitions nocturnes dès le stade de l'enquête préliminaire ou en cas de procédure de flagrance.

la sonorisation des lieux privés et la captation à distance de données informatiques. Nous avons renforcé les règles de contrôle d'identité en autorisant la retenue de quatre heures de la personne contrôlée.

lequel va créer de nouveaux pouvoirs de police permanents dans le droit commun, afin de répondre à l'exigence impérieuse de sécurité et de protection de nos concitoyens. Certaines de ces dispositions sont inspirées de l'état d'urgence : l'instauration de périmètres de protection, la fermeture administrative des lieux de culte, la création de mesures individuelles de surveillance, ainsi que les visites de domiciles et les saisies. Avec ce texte, l'État sera doté de moyens forts au profit de nos forces de sécurité et de nos services de renseignement.

présider. En limitant le champ d'application de cette loi aux fins de prévenir des actes terroristes, notre législation de droit commun diffère de l'état d'urgence, lequel peut être instauré pour tout motif de sécurité publique. au texte cette fameuse « clause d'autodestruction » imposant une limite de validité, au 31 décembre 2020, des quatre mesures emblématiques du texte, le Sénat a programmé l'obsolescence d'un droit nécessaire à un moment donné de l'histoire. Enfin, en accroissant le contrôle parlementaire au moyen d'une information sans délai du Parlement ainsi que de la remise annuelle au Parlement d'un rapport détaillé sur l'application des dispositions les plus attentatoires aux libertés, cette loi renforce notre démocratie. En renforçant le contrôle du juge pour la mise en oeuvre des dispositions importantes, nous rappelons le rôle primordial de garant des libertés individuelles du juge judiciaire. En introduisant des mesures de prévention au respect du droit à la vie privée et à la protection des données personnelles, comme l'accès indirect aux fichiers PNR- -ou la limitation des des contrôles aux frontières, le Sénat s'impose comme le gardien d'un équilibre démocratique précieux dans un État de droit auquel nous sommes attachés, sans pour autant abandonner des outils absolument nécessaires pour lutter contre le fléau du terrorisme. Vous l'avez compris, notre groupe votera bien sûr ce texte.

aujourd'hui. Mais sera-t-il suffisant pour venir à bout du terrorisme aux mille entailles qui atteint aujourd'hui l'Europe ? Je n'en suis pas certaine. En effet, nous sommes dans une guerre de l'obus et du blindage. Nous sommes dans la réaction systématique. Aujourd'hui, nous multiplions les contrôles,

nous multiplions -les ingérences dans la vie privée, mais vous privez, madame la ministre, les communes d'un élément essentiel en matière de contrôle de leur population, à savoir l'élaboration des cartes nationales d'identité, ainsi que les autorisations de sortie du territoire, et vous vous opposez systématiquement aux demandes de nos collègues alsaciens d'étendre à tout le territoire

Vous le comprenez bien, tous les imams détachés des pays d'origine constituent autant de risques. Certes, le Maroc est l'islam du juste milieu, mais vous avez bien vu la part jouée par cet imam marocain dans l'attentat de Barcelone. Qu'en serait-il aujourd'hui si une chose pareille arrivait en France ? absolument avancer sur ces éléments. Oui, je partage les propos d'Éliane Assassi : il faut absolument travailler sur le volet de la prévention. Que va-t-on faire des 12 000 personnes radicalisées signalées à l'UCLAT,

en hommes et en matériels. Il faut absolument se saisir de la question de la lutte contre la radicalisation et de la prévention, sauf à continuer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

adopté définitivement. Voici le résultat du scrutin pour l'élection de six juges titulaires à la Cour de justice de la République et de leurs six juges suppléants Nombre de votants : 311 Suffrages exprimés : 304 Majorité absolue des suffrages exprimés : 153 Bulletins blancs : 4 Bulletins nuls : 3 Ont obtenu M. Arnaud de Belenet, titulaire, et M. Bernard Cazeau, suppléant, 304 voix ; M. François-Noël Buffet, titulaire, et Mme Catherine Troendlé, suppléante, 304 voix Mme Agnès Canayer, titulaire, et Mme Brigitte Lherbier, suppléante, 304 voix ; M. Yves Détraigne, titulaire, et Mme Françoise Férat, suppléante, 304 voix M. François Pillet, titulaire, et Mme Catherine Di Folco, suppléante, 304 voix ; Mme Laurence Rossignol, suppléante, 304 voix ; Mme Laurence Rossignol, titulaire, et M. Jean-Luc Fichet, suppléant, 304 voix. Ces candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, ils sont proclamés juges à la Cour de justice de la République. Mmes et MM. les juges titulaires et Mmes et MM. les juges suppléants à la Cour de justice de la République vont être appelés à prêter, devant le Sénat, le serment prévu par l'article 2 de la loi organique du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République. Je vais donner lecture de la formule du serment. Il sera procédé ensuite à l'appel nominal de Mmes et MM. les juges titulaires, puis à l'appel nominal de Mmes et MM. les juges suppléants. Je les prie de bien vouloir se lever à l'appel de leur nom et de répondre, en levant la main droite, par les mots : « Je le jure. » Voici la formule du serment : « Je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions,

Acte est donné par le Sénat du serment qui vient d'être prêté devant lui. Mme Agnès Canayer, qui n'a pu assister à la séance d'aujourd'hui, sera appelée ultérieurement à prêter serment devant le Sénat.